monsieur le président.

La fixation du rythme annuel d'alimentation et des plafonds des droits liés au compte personnel de formation des agents publics relèvent du domaine réglementaire. Dans sa décision sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Conseil constitutionnel a validé, pour le secteur privé, le transfert au niveau réglementaire de la fixation

Enfin, recourir aux ordonnances, alors même que le présent projet de loi vise une réforme d'ensemble et en profondeur de la fonction publique, nous semble contradictoire. Sur le fond, cet article va favoriser l'intégration des logiques du dès la formation initiale des fonctionnaires, ainsi que dans leur formation continue. De plus, en l'état, les objectifs sont trop flous pour que nous signions un chèque en blanc au Gouvernement. Que signifie concrètement la réforme des voies d'accès ? Le système universel du recrutement par concours sera-t-il mis à mal ? Quelle place attribuer aux contractuels et aux intervenants privés ? Nous rappelons à cet égard que l'égalité d'accès aux concours de la fonction publique est un principe général du droit depuis le fameux arrêt du Conseil d'État de 1954. Nous nous opposons donc à la philosophie même de cet article, qui met sur le même plan la mobilité entre les trois fonctions publiques et la mobilité vers le privé. Pour résumer, alors que de réels problèmes d'inégalité d'accès, de manque de formation

ailleurs, en pleine polémique sur la suppression de l'ENA, annoncée par le Président de la République, les questions de formation, de la base au sommet de l'échelle de la fonction publique, méritent plus qu'une ordonnance : un débat public au Parlement.

Nous avons choisi la seconde option et fait des choix extrêmement forts, en refusant toute fusion d'écoles dans le cadre de l'ordonnance et toute réforme à l'aveugle du financement du CNFPT, en précisant nos attentes concernant la diversification de la haute fonction publique, notamment pour développer les classes préparatoires intégrées, et en encourageant l'État à mieux gérer les parcours de carrière de ses agents. Par ailleurs, madame Assassi,

Assassi, le concours restera la pierre angulaire de l'accès aux écoles de la fonction publique, quel que soit le niveau de qualification. Nous souhaitons que le concours reste le mode de recrutement des agents titulaires. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous avons ouvert une concertation

Le scrutin est ouvert.

secrétaire d'État. Il s'agit de rétablir la rédaction que l'Assemblée nationale avait adoptée, à la demande du Gouvernement, s'agissant à la fois de la coordination des écoles et des perspectives à ouvrir en matière de réforme de la haute fonction publique.

le texte adopté à l'Assemblée nationale. Cette rédaction nous semble beaucoup trop large pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui impose de connaître les finalités et le périmètre de l'ordonnance. Avec le texte du Gouvernement, toutes les écoles de service public de catégorie A pourraient être concernées, tout comme, d'ailleurs, une réforme du CNFPT. La rédaction de la commission rend service au Gouvernement, en réalité, en réduisant le risque de censure si ce texte devait être déféré au Conseil constitutionnel après son adoption. En outre, le texte du Sénat ne gêne en rien la mission Thiriez : nous nous sommes d'ailleurs inspirés de sa lettre de mission pour l'écrire et nous avons rencontré M.

services publics. Or la seule référence aux activités professionnelles conduit finalement à faire bénéficier de cette troisième voie d'accès des personnes dont le profil, les études et les parcours de vie ne sont pas fondamentalement différents

titre de ce concours. Le troisième concours a été créé pour diversifier les profils de recrutement de cette école. Le supprimer pénaliserait les salariés de grands groupes, mais également les responsables associatifs, ce qui n'est sans doute pas la volonté du groupe CRCE.

des fonctionnaires de police ou de gendarmerie nationale qui intègrent le cadre d'emploi de la filière de la police municipale. Le Gouvernement partage l'avis et l'objectif de la commission. Néanmoins, nous pensons préférable de modifier la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique plutôt que le code de la sécurité intérieure, qui comporte d'ores et déjà une disposition permettant, pour toutes les filières, de tenir compte des formations professionnelles antérieures pour réduire la durée de la formation obligatoire dispensée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. La rédaction vise précisément la filière de la police municipale. Les décrets statutaires des différents cadres d'emploi de cette filière pourront ainsi être modifiés pour préciser les conditions dans lesquelles la durée des formations pourra être réduite, en particulier pour les fonctionnaires de police ou de gendarmerie nationale qui voudraient intégrer la police municipale.

pas dans le code de la sécurité intérieure, mais dans la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Sur le fond, la rédaction proposée publique territoriale. Sur le fond, la rédaction proposée par le Gouvernement ne nous semble pas équivalente à celle que nous avons introduite en commission. Elle conduit en effet à moduler la durée de formation des agents de police municipale en fonction non pas de l'expérience professionnelle antérieure, mais des formations professionnelles et des bilans de compétences effectués par l'agent au cours de sa carrière. la loi du 12 juillet 1984 ne comporte que des dispositions générales. Il apparaît peu opportun de commencer à y intégrer des dispositions spécifiques à un cadre d'emploi, quand il s'agit de la fonction publique territoriale. Notons d'ailleurs

d'orthoptiste et d'orthophoniste, en raison de la création d'un statut d'apprenti pour les auxiliaires médicaux. Le recours à cette solution sacrifierait la qualité des soins, la formation des étudiants, et pourrait entraîner des dérives. La formation se ferait « sur le tas

En effet, l'article 22 A vise clairement quatre filières : les masso-kinésithérapeutes, les orthoptistes, les pédicures-podologues et les orthophonistes. La question de sa pertinence se pose, dès lors qu'il confère aux employeurs hospitaliers la possibilité d'avoir recours à des apprentis. Dans certains cas, comme celui des orthophonistes, paraît particulièrement inadapté, dès lors qu'il est déjà difficile, pour les étudiants orthophonistes, de trouver des maîtres de stage disposés à l'accueillir. De façon globale, cet article laisse craindre un recours dévoyé à l'apprentissage, destiné à combler les vacances de postes. Quel est

Il suscite l'inquiétude chez certains professionnels, notamment les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes. Il faut dire que la méthode suivie par le Gouvernement n'est pas idéale : l'article a été introduit à l'Assemblée nationale, sans étude d'impact et sans véritable concertation avec les professionnels, alors même que le Sénat

Il faut donc mieux articuler le code du travail, qui autorise l'apprentissage, et le code de la santé publique, qui interdit l'exercice illégal de la profession. Développer l'apprentissage dans la fonction publique hospitalière semble nécessiter de tels ajustements. Le Gouvernement doit toutefois rassurer les professionnels sur la formation des apprentis et apporter les moyens nécessaires.

Les pratiques et les actes qu'ils sont appelés à commettre doivent être encadrés et proportionnés aux compétences qu'ils ont acquises. L'avis est défavorable.

Les étudiants et étudiantes en orthophonie préparent leur diplôme uniquement au sein de l'université. Leurs frais de scolarité sont limités aux frais d'inscription à l'université. Actuellement, vingt universités proposent cette formation théorique, mais aussi pratique, des stages réalisés auprès de maîtres de stage non rémunérés. La formation d'orthophoniste n'existe pas sous la forme de l'apprentissage. Il n'y a donc pas de raison d'étendre le statut de l'apprentissage qui existe éventuellement dans d'autres professions de santé. De plus, profession connaît une pénurie au sein de la fonction publique hospitalière et des structures médico-sociales, du fait d'un statut et de salaires peu attractifs. Il serait donc inenvisageable, pour des apprentis en orthophonie, de trouver des maîtres d'apprentissage conformément à l'article L. 6223-5 du code du travail,

dans la formation initiale des futurs orthophonistes. La parole

commission ? L'article 22 A ouvre la porte au développement de l'apprentissage pour la profession d'orthophoniste. Cette profession s'est fortement mobilisée pour contester cette disposition. L'apprentissage n'existe pas chez les orthophonistes, mais c'est peut-être l'occasion d'évoluer en ce sens Il revient au Gouvernement de mieux consulter les professionnels sur les évolutions envisagées, notamment en matière de formation. L'adoption de ces amendements permettait, au moins, de laisser ouverte la discussion sur cet article, qui ne fait pas l'unanimité, jusqu'à la commission mixte paritaire. Nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

CNFPT soutienne le développement de l'apprentissage en le finançant à 75 %, tel que c'était prévu initialement, ou à 20 %, tel que l'amendement adopté en commission le prévoit, n'est pas une mauvaise idée, à condition que les dépenses supplémentaires que cela implique soient compensées par une augmentation de ses moyens. En l'absence d'une telle compensation, le CNFPT, dont la mission de formation des agents publics territoriaux est essentielle, serait obligé de répercuter ces dépenses supplémentaires sur des formations qu'il propose actuellement. Cela reviendrait, en quelque sorte, déshabiller Pierre pour habiller Paul, ce qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux liés au soutien à l'apprentissage dans la fonction publique et à la formation continue des fonctionnaires et des agents de la fonction publique.

dont l'objectif était de contraindre le CNFPT à verser aux centres de formation d'apprentis une contribution ne pouvant, en tout état de cause, être inférieure à 75 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et certains de leurs établissements publics.

des fonctionnaires ou les possibilités d'ouverture de postes en apprentissage dans les collectivités, au sein des services publics. Vous le savez, mes chers collègues, l'apprentissage et l'alternance sont au centre de mes préoccupations. J'ai d'ailleurs posé une question d'actualité au Gouvernement sur que la solution proposée n'est pas viable ni envisageable en pratique. Demander au CNFPT de financer les frais de formation des apprentis, sans lui apporter aucune recette supplémentaire, aura inévitablement des répercussions importantes sur son fonctionnement et sa capacité de financement des formations des agents territoriaux. Il nous faut effectivement trouver des solutions pérennes au problème du financement de l'apprentissage, mais sûrement pas en remettant en cause le droit à la formation des agents territoriaux. Il est par conséquent nécessaire de mettre en oeuvre une concertation sur ce sujet entre le Gouvernement, le CNFPT,

de la commission ? L'article 22 B, introduit à l'Assemblée nationale, vise à trouver des solutions pour le financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Les apprentis des collectivités sont en effet les grands oubliés de la loi Pénicaud du 5 septembre 2018. Dépouillées de leur compétence en matière d'apprentissage, les régions ne participeront plus au financement de leur formation. La commission a proposé une solution de compromis pour maintenir les finances du CNFPT, soient pris en charge à hauteur de 30 % par l'État, soit 23 millions d'euros, de 20 % par le CNFPT, soit 15 millions d'euros, et de 50 % par les employeurs territoriaux. Le CNFPT bénéficierait, en outre, d'une adaptation de ses flux financiers avec les centres de gestion. Le Gouvernement et Mme Françoise Gatel proposent d'autres solutions, que nous allons examiner au travers des amendements suivants. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement qui revient sur l'effort de compromis mené de part et d'autre.

les régions exerçaient la compétence en matière d'apprentissage, finançaient les CFA et les frais de formation des apprentis. Certaines régions finançaient

cette forme d'incongruité qui consistait à financer une activité de formation publique avec de l'argent privé. Aujourd'hui, nous devons trouver une solution pour permettre un meilleur financement de l'apprentissage.

en application de la loi de 2016 qui lui donne compétence en matière d'apprentissage, et 30 % par un prélèvement sur recettes de l'État. Le Gouvernement ne peut agréer cette proposition de la commission des lois. Nous considérons que les employeurs territoriaux et les organismes qui les fédèrent sont compétents en matière de formation des agents territoriaux, de même que l'État est compétent pour la formation de ses agents. J'ai J'ai dit sous forme de boutade, à l'occasion d'une autre discussion, que si l'on entérinait le principe d'un financement de l'apprentissage dans les collectivités par un fonds d'État, il faudrait peut-être envisager un financement de la formation continue des agents de l'État par un fonds de concours des collectivités, pour que chacun puisse s'y retrouver

ne pourra faire l'économie d'une réflexion sur les charges de gestion du CNFPT, qui s'élèvent à 12 % de ses recettes, soit 40 millions d'euros. Ce montant est important. Un certain nombre des dispositions adoptées par votre commission des lois, notamment en matière de réorganisation territoriale, nous semblent devoir concourir à cette

le Premier ministre a lancé une mobilisation générale pour l'emploi, en particulier pour le soutien à l'apprentissage. J'imagine que sur l'ensemble des travées de la Haute Assemblée, nous partageons cet objectif.

pour que l'apprentissage puisse être financé de manière raisonnable, sans prélèvement supplémentaire sur les collectivités et sans ponction sur les deniers de l'État. La parole

la commission est peut-être le moins mauvais. Pour notre part, nous avions déposé un amendement qui a subi les foudres de l'article 40 parce que nous souhaitions

on commence à voir apparaître des déserts administratifs. Les petites collectivités qui emploient et forment dans de bonnes conditions les apprentis ont aujourd'hui beaucoup de mal

commission ? Dans le secteur public, la rémunération de l'apprenti dépend de deux paramètres : son âge et le type de formation suivie. La rémunération des apprentis de niveau post-bac est de 10 % à 20 % supérieure à celle des autres apprentis. Cette situation soulève aujourd'hui une difficulté, car les collectivités territoriales et l'État recrutent de plus en plus d'apprentis post-bac, ce qui accroît les coûts de recrutement. L'amendement n° 410 du Gouvernement tend à supprimer cette bonification pour les apprentis post-bac, alignant le secteur public sur le secteur privé. L'employeur pourra toujours verser des primes aux apprentis afin de valoriser les profils les plus intéressants. L'avis de la commission est favorable.

est la principale conclusion formulée dans le rapport d'information de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication intitulé « Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation », publié en 2018. Ses préconisations portent sur la sensibilisation au numérique et l'accompagnement des agents publics des collectivités territoriales, le renforcement de la formation des délégués académiques dans le même domaine et le recours à des moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats. Cet amendement, qui s'inscrit dans le prolongement d'une disposition introduite dans le projet de loi pour une école de la confiance, vise à renforcer et à préciser les axes prioritaires du volet numérique de la formation initiale et continue des enseignants. En effet, seule la formation de l'ensemble des acteurs, y compris ceux des administrations et les agents publics, pourra permettre à la France et à l'Union européenne d'assurer leur souveraineté numérique. Les révélations sur les écoutes de la, la NSA, ont montré que les fonctionnaires étaient des cibles privilégiées. C'est pourquoi, afin de préserver notre souveraineté et la neutralité du service public face aux Gafam, il est essentiel de les sensibiliser à l'utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.

Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, pour diversifier aussi les parcours professionnels des agents publics, nous proposons de déployer à titre expérimental, dans la fonction publique d'État, un dispositif de mécénat de compétences auprès d'associations déclarées d'intérêt général. Ce dispositif prendrait la forme d'une mise à disposition dérogatoire au droit commun, en tant qu'elle pourrait intervenir auprès d'associations relevant de l'une des catégories d'intérêt général mentionnées à l'article 238 du code général des impôts. Il ne pourrait donner lieu à un remboursement, d'où l'appellation de mécénat. Compte tenu de son inscription dans une logique de projet, cette mise à disposition ne pourrait excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite de trois

de cette mise à disposition, pour la conduite ou la mise en oeuvre d'un projet pour lequel les compétences professionnelles des agents concernés peuvent être utiles à l'association,

supprimer l'article. Les militaires bénéficient déjà d'un droit à la mobilité temporaire en dehors du service. Cependant, le législateur, reconnaissant le caractère central et régalien de la défense nationale, a voulu instaurer des garde-fous

poser trop de difficultés, même si la majeure partie de ces entreprises peuvent déjà accueillir des militaires au titre de leurs activités de défense. Plus problématique est le cas des entreprises privées de surveillance et de sécurité : les deux métiers sont profondément différents. Enfin, le cas des sociétés militaires privées Notre groupe souligne depuis plusieurs années les dérives de ces sociétés de mercenariat, dont la reconnaissance législative par la France, en 2014, interroge au regard du droit international, alors même que le Conseil de sécurité de l'ONU a pointé, en février dernier, le rôle des mercenaires dans l'insécurité dans l'insécurité en Afrique. Notre groupe dénonce l'abandon progressif de missions par les armées régulières au profit de sociétés privées agissant en toute impunité.

La crainte d'une dérégulation avancée par les auteurs de cet amendement ne me semble pas fondée. En tant que militaires en activité, les personnes concernées demeureraient soumises aux dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la défense, qui proscrit, par principe, l'exercice de toute activité privée lucrative, à l'exception des activités prévues

par les collectivités locales dans le cas où une réintégration de l'agent en surnombre ne pourrait être compensée.

soulèvent deux difficultés pour les collectivités frontalières : d'une part, il leur faut gérer ces départs et réorganiser les services ; d'autre part, il leur faut parfois prendre en charge l'allocation de retour à l'emploi, sur la base d'un salaire suisse. Il s'agit sans doute d'un amendement d'appel,

peut s'opérer d'un cadre d'emploi à un autre au sein d'une même collectivité, ou dans une autre collectivité. Lorsque le fonctionnaire change de collectivité en conservant le même cadre d'emploi, il s'agit d'une simple mutation, qui ne s'opère pas par la voie du détachement. C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article. Quel est

Il a pour objet d'autoriser le détachement d'un fonctionnaire territorial sur plusieurs emplois à temps non complet. Je reconnais qu'une telle situation peut provoquer des difficultés de gestion. En revanche, contrairement à ce qui est écrit dans l'objet de l'amendement, je ne vois pas ce qui empêche le détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi relevant du même cadre d'emploi auprès d'un autre employeur.

de déroger au principe d'interdiction du double détachement dans le cas particulier où le fonctionnaire désire continuer à exercer le même emploi fonctionnel qu'avant sa promotion.

de la commission ? Sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Grand, la commission a supprimé l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein d'une commune membre de l'EPCI. Cette incompatibilité crée en effet une différence de traitement entre les agents de l'EPCI, qui peuvent se présenter aux élections municipales, et ceux des communes membres, qui ne peuvent pas devenir conseillers communautaires. Le Gouvernement a lui-même reconnu le problème, dans une réponse écrite publiée le 6 décembre 2018. Cette disposition a bien un lien avec le texte, car elle renforce les droits civiques des agents publics.

À l'occasion de nos discussions avec les associations d'élus et les représentants des employeurs territoriaux, nous avions évoqué l'éventualité d'élargir les possibilités de primo-recrutement en CDI dans la fonction publique territoriale. Les employeurs territoriaux nous avaient alors indiqué ne pas y être favorables : ils préféraient s'en tenir à des modes de recrutement statutaires ou à des recrutements contractuels plus classiques, à durée déterminée. Votre commission a fait le choix d'élargir la possibilité de procéder à des primo-recrutements en CDI dans la fonction publique territoriale. Le Gouvernement, fidèle aux engagements pris devant les employeurs territoriaux, souhaite revenir sur cette disposition.

La portabilité du CDI, je le rappelle, n'est pas un droit pour l'agent, mais une faculté, pour l'employeur qui recrute un agent contractuel sur certains emplois, de lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée si l'agent était précédemment employé en CDI. La portabilité est donc une dérogation à la règle qui interdit traditionnellement de recruter un agent contractuel de droit public en CDI. Or cette règle n'existe déjà plus dans la fonction publique hospitalière. projet de loi prévoit en outre de supprimer la plupart des obstacles au recrutement initial en CDI dans la fonction publique de l'État, précisément sur les emplois concernés par la portabilité. Par conséquent, la portabilité du CDI n'a plus de sens dans ces deux versants de la fonction publique, qu'elle s'applique au sein d'un même versant ou d'un versant à l'autre. Le projet de loi ne maintenait l'interdiction du primo-recrutement en CDI que dans la fonction publique territoriale. La commission des lois était donc confrontée au choix suivant : soit ne maintenir les dispositions relatives à la portabilité du CDI que dans la fonction publique territoriale, soit supprimer, dans celle-ci comme dans les deux autres versants, les obstacles au primo-recrutement en CDI. C'est la seconde option que nous avons Je précise qu'il ne s'agit pas d'élargir les conditions de recrutement au contrat. Il nous a simplement semblé que, lorsque le recrutement d'un agent contractuel est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service et qu'il a été impossible de pourvoir l'emploi en recrutant un fonctionnaire, il n'y a pas de raison d'interdire à l'employeur territorial d'embaucher directement en CDI. Ce n'est pas en entretenant la précarité parmi les agents contractuels que l'on renforcera l'attractivité des concours de la fonction publique territoriale. C'est pourquoi la

au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. C'est un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Il y a déjà, dans la fonction publique, plusieurs dispositifs qui équivalent à des formes de Le dispositif proposé ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sous contrat, ni ceux qui ont droit à une pension de retrait à taux plein. le secrétaire d'État, c'est que vous prévoyez le remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle, sous certaines conditions, en cas de retour dans l'emploi public.

Gouvernement est de fluidifier les carrières et les départs vers le secteur privé. Il restreint en fait les perspectives de carrière des fonctionnaires et facilite leur départ. La rupture conventionnelle est introduite à titre expérimental, pour une durée de six ans, avec un point d'étape au bout de cinq ans, ce qui ne garantit en rien la transparence du dispositif. Elle ouvre droit à une indemnité remboursable en cas de retour dans l'administration d'origine. La version initiale du texte prévoyait ce remboursement en cas de retour dans les trois ans ; la majorité de l'Assemblée nationale a porté ce délai Pour s'assurer du respect des conditions légales et du libre consentement des parties, la rupture conventionnelle fera l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Ce point pose question, dans la mesure où l'administration est partie prenante à la

le Gouvernement se dote en fait d'un moyen supplémentaire pour atteindre ses objectifs de diminution de l'emploi public. Il s'agit, ni plus ni moins, d'un instrument de gestion des effectifs. Enfin, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, on peut s'étonner que l'étude d'impact ait fait l'impasse sur les conséquences financières de ces articles pour les employeurs.

? La commission n'est pas favorable à la suppression de cet article qui, en plus d'instituer une rupture conventionnelle dans le secteur public, étend le bénéfice de l'assurance chômage à de nouvelles catégories d'agents publics. Elle a donc émis

S'ils sont titulaires, ils peuvent faire valoir, dans des conditions assez restrictives, le droit à une indemnité de départ volontaire, mais celle-ci n'est absolument pas accompagnée d'une allocation de retour à l'emploi.

Cet amendement a pour objet de rétablir la précision selon laquelle la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. C'est ce que l'on appelle la liberté de consentement. Cette garantie figure dans le code du travail pour les salariés de droit privé. Il nous apparaît utile de l'inscrire dans la loi pour les agents publics concernés.

lors du comité interministériel de la transformation publique du 1 février 2018, l'article 26 prévoit l'expérimentation d'un dispositif de rupture conventionnelle visant, aux termes de l'étude d'impact, à favoriser la fluidité des carrières entre l'emploi public et le secteur privé. Lors de l'examen de la proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires, nous avions constaté la grande faiblesse de l'information disponible concernant les cas définitifs de sortie de la fonction publique, les personnes concernées n'ayant pas intérêt à régulariser leur situation. Si l'on peut souscrire à l'objectif de rénovation du cadre de sortie de l'emploi public, il est à craindre que l'introduction d'un tel dispositif donne lieu à d'importantes négociations dans tous les versants de la fonction publique. Comme le souligne l'étude d'impact, le nombre à venir de ruptures conventionnelles, qui constituent un nouveau cas de sortie de la fonction publique, est impossible à estimer ». Dans le secteur privé, la création de la rupture conventionnelle répondait à un besoin d'apaisement des relations professionnelles en cas de rupture anticipée du contrat de travail de diminuer le recours aux abandons de poste. Du fait du coût de l'indemnité versée par l'employeur en cas de rupture conventionnelle, ce dispositif n'a pas tenu toutes ses promesses, d'où l'idée de créer un droit à la démission.

Si l'introduction d'une possibilité de rupture conventionnelle rencontrait un grand succès, elle pourrait donc considérablement déstabiliser certains services. Afin de prévenir ce risque, nous proposons d'inscrire dans la loi que la préservation de l'intérêt général peut fonder une décision de refus de rupture conventionnelle. Quel

considérant l'intérêt du service. C'est sans doute ce qu'aurait explicité le juge, mais cela va mieux en l'écrivant, car cela garantit un très large pouvoir d'appréciation à l'employeur.

ce dernier, car l'administration qui versera l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas nécessairement celle qui, le cas échéant, aura droit au remboursement de la pantoufle. Je rappelle que les fonctionnaires qui n'ont pas honoré leur engagement de servir sont, en tout état de cause, tenus de rembourser les sommes perçues, au prorata du temps de service restant à accomplir.

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à rétablir l'homologation de la convention de rupture conventionnelle par l'autorité administrative, supprimée en commission. Qu'une autorité administrative homologue une convention passée par une autre autorité administrative est déjà assez curieux. Pour contrôler l'action de l'administration, il existe une institution qui a fait ses preuves, à savoir la juridiction administrative. Qui plus est, il serait inacceptable qu'une convention de rupture conventionnelle passée par un employeur public territorial soit soumise à l'homologation d'une d'une autorité administrative de l'État, comme le préfet. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler, mes chers collègues, que, depuis la loi du 2 mars 1982, les actes des autorités locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification et, pour certaines catégories d'entre eux, leur transmission au représentant de l'État. Les collectivités n'ont plus à demander à M. le préfet son accord pour prendre des décisions ou conclure des conventions. Depuis 2009, la révocation ou le licenciement d'un fonctionnaire territorial ne sont même plus soumis au contrôle de légalité. La commission émet donc un avis très défavorable

comme la loi le prévoit, de consacrer le rôle du conseiller syndical, que nous avons introduit après la publication de l'avant-projet de loi à la demande des organisations syndicales. Il précisera également les conditions dans lesquelles les employeurs publics seront amenés à participer au financement de l'allocation de retour à l'emploi. Nous fixons donc des garanties. Nous n'en sommes pas encore au stade

qui n'ont pas rempli l'intégralité de leurs obligations de service ne leur permette d'échapper au remboursement de leur formation. C'est un point vraiment essentiel. Les grandes écoles coûtent cher, tout comme la formation qui est à la charge de l'État. Les fonctionnaires qui sont recrutés par ce biais bénéficient d'un enseignement de très grande qualité, onéreux donc pour la collectivité.

au respect de l'engagement pris, soit au remboursement de la pantoufle. Le sous-amendement vise également à supprimer le II de l'amendement, car nous tenons à maintenir les dispositions selon lesquelles un fonctionnaire recruté par un autre employeur du même versant dans les années qui suivent une rupture conventionnelle doit rembourser l'indemnité perçue.

en cas de retour au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement avec lequel il avait convenu d'une rupture conventionnelle. Outre le fait que le délai nous paraît excessivement long, l'articulation d'un délai de six ans avec le caractère expérimental du dispositif pour une durée de cinq années pose question. Il est donc proposé d'en rester au délai de trois Marie. Il s'agit de mieux circonscrire, pour la fonction publique de l'État, le périmètre auquel s'applique l'obligation de remboursement des sommes perçues lors de la rupture conventionnelle en cas de retour. en cas de retour. Ce périmètre nous paraît excessivement large, puisqu'il englobe sans distinction tous les emplois au sein de la fonction publique de l'État, ce qui crée une différence de traitement avec les fonctions publiques territoriale et hospitalière pour lesquelles le texte n'applique l'obligation de remboursement qu'en cas de retour dans la même collectivité ou dans le même établissement de santé. Par équité entre les agents des trois versants, nous proposons de circonscrire l'obligation de remboursement pour les agents de la fonction publique de l'État en cas de retour au sein de l'administration de l'État ou de l'établissement public d'État avec lequel il a été convenu une rupture conventionnelle.

l'amendement n° 160 rectifié, qui vise à réduire de six à trois ans le délai de latence pendant lequel un agent qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle ne peut être recruté dans le secteur public sans avoir à rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue.

Le projet de loi prévoit qu'un agent qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle ne puisse être recruté dans le secteur public, dans un délai de six ans, sans avoir à rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue. perçue. Or le périmètre de cette interdiction n'est pas le même dans les trois versants. Dans la fonction publique territoriale, l'agent aurait l'interdiction d'être recruté par la même collectivité territoriale ou par un établissement public qui en relève, sauf à rembourser son indemnité. Nous proposerons de corriger l'oubli du cas où l'administration territoriale d'origine est un établissement public. Dans la fonction publique hospitalière, l'agent aurait l'interdiction d'être recruté par le même établissement. Dans la fonction publique de l'État, en revanche, il aurait l'interdiction d'être recruté par n'importe quelle administration d'État. Il faut avouer qu'il y a là un défaut de parallélisme. Toutefois, il semblerait plus opportun et plus légitime d'élargir le périmètre de l'interdiction dans les trois versants que de le réduire pour la Les textes qui régissent l'indemnité de départ volontaire prévoient, quant à eux, une obligation de remboursement dans le cas où l'agent est recruté dans n'importe lequel des trois versants dans un délai de cinq ans. Encore une fois, il faut faire attention aux effets d'aubaine, car ce sont les employeurs publics, donc les contribuables, qui paieront. Par conséquent, la

en plus d'autorisations spéciales d'absence et d'un crédit de temps syndical, de diverses garanties en termes d'avancement et de rémunération notamment, ne sont pas assimilables aux salariés protégés. Ils ne disposent par exemple d'aucune garantie particulière en matière de discipline ou de licenciement. Par conséquent, la commission demande le

La période de deux ans proposée est trop courte. L'amendement n° 416 tend à clarifier les droits à l'assurance chômage des agents contractuels de droit public, dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage de droit commun. Il s'agit à la fois de sécuriser les droits à l'allocation chômage des agents contractuels, alors que les textes actuels rendent possibles des interprétations divergentes, et de garantir l'équité entre ces agents contractuels et ceux dont l'employeur est resté en auto-assurance chômage, en prévoyant que les droits à l'allocation chômage des premiers puissent être identiques à ceux des seconds.

que le Premier ministre transmet avant toute négociation des accords relatifs à l'assurance chômage. À notre sens, il n'y a aucune raison de consulter le CCFP sur des accords qui concernent le seul secteur privé du fait du périmètre du document de cadrage.

au lieu d'être leurs propres assureurs. Dans ce cas, ils acquittent des cotisations sur les rémunérations versées à ces agents, et c'est l'Unédic qui, le cas échéant, prend en charge l'allocation chômage. Il en va notamment ainsi des employeurs publics territoriaux exclusivement pour leurs agents contractuels. Par l'amendement Par l'amendement n° 416, le Gouvernement veut garantir aux agents concernés le droit à l'assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents couverts par l'auto-assurance, c'est-à-dire en cas de privation involontaire d'emploi, à la suite d'une rupture conventionnelle ou d'une démission ouvrant droit à indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration. Une telle disposition ne nous paraît pas nécessaire, car ces agents sont déjà inclus parmi ceux qui sont mentionnés à l'alinéa 15 de l'article 26. Néanmoins,

sont définies par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage, s'appliquent aux employeurs et agents publics, alors même qu'ils ne participent pas à leur élaboration. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les employeurs publics sont, en règle générale, leurs propres assureurs en la matière : ils assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage de leurs agents au lieu d'être affiliés au régime d'assurance chômage. L'extension du bénéfice de l'assurance chômage aux agents publics bénéficiant d'une rupture conventionnelle et à certains agents publics démissionnaires pourrait peser lourdement sur les budgets publics. C'est pourquoi la commission des lois a estimé nécessaire que les représentants des employeurs et des agents de la fonction publique

sauf dans le cas où la collectivité a été victime d'un acte délictuel de la part de l'agent révoqué : vol, détournement de fonds ... En effet, la collectivité victime se trouve alors dans la situation incompréhensible, notamment pour le contribuable, de devoir indemniser l'auteur de son préjudice.

? Ce sont des sujets assez délicats et complexes. Nos collègues proposent de priver du droit à l'assurance chômage les fonctionnaires révoqués « pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive Je conçois volontiers que les employeurs publics en auto-assurance aient du mal à comprendre qu'ils doivent supporter le coût de l'allocation d'assurance chômage versée à des fonctionnaires révoqués dans ces conditions.

même nature. Par ailleurs, le droit français a toujours considéré la privation d'emploi pour motif disciplinaire comme un cas de privation involontaire d'emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Un salarié de droit privé licencié pour faute lourde a droit à l'assurance chômage je vous renvoie à l'article 2 du règlement général annexé à la convention nationale d'assurance chômage. L'équité entre le secteur public et le secteur privé doit s'appliquer dans les deux sens. Enfin, la privation du droit à l'assurance chômage pourrait être considérée comme une peine complémentaire automatique, contraire au principe constitutionnel d'individualisation des peines. Si le fonctionnaire révoqué ou le salarié licencié pour faute lourde ont droit à l'assurance chômage, ils n'ont évidemment droit à aucune indemnité liée à la perte de leur emploi.

rapporteur. Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé.

jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une nouvelle affectation. Pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en contrat Dès lors, lorsqu'un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l'agent contractuel qui l'a remplacé doit être reclassé ou licencié, et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi. Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales, notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d'une commune soit mis en disponibilité pendant des années et des années pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement au poste, car aucun agent suffisamment qualifié n'accepte d'être recruté sur contrat, au risque d'être licencié dès que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l'employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s'expose à devoir assumer la charge financière d'un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité sollicitera sa réintégration. Pour mettre fin à cette situation inextricable, le présent amendement vise, d'une part, à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit pour raisons familiales, selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif- autre motif- élever un enfant âgé de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, etc. part, à faire en sorte qu'un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d'office que si la durée de la disponibilité de droit n'a pas excédé trois ans. Au-delà de cette période, l'agent conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d'origine. Ces dispositions entreraient en vigueur le 1 janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.

de l'intention de favoriser les mobilités pour faciliter et anticiper les transformations professionnelles. En ne ciblant que les agents dont l'emploi est supprimé, cet article est de nature à et rend le travail des directions des ressources humaines plus compliqué. Tout agent faisant partie d'un service ou d'une direction restructuré doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement à la transition professionnelle. En outre, les dispositifs de prise en charge des agents ayant perdu leur emploi mis en oeuvre par les centres de gestion et le CNFPT dans la fonction publique territoriale ne couvrent qu'une partie de l'accompagnement en transition professionnelle.

à ceux dont l'emploi est supprimé, comme le prévoit le projet de loi, ainsi qu'à tout fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui, à cette occasion, démissionne de bénéficier d'une indemnité de départ volontaire,

tant des objectifs politiques que des limites propres au contenu de cet article. Tout d'abord, ce nouvel aménagement de l'accompagnement des agents dont l'emploi est supprimé est indissociable des vastes plans de suppressions de postes d'agents publics. Les conditions ont déjà été mises

dans la fonction publique, auxquelles, vous le savez, mes chers collègues, nous nous opposons fortement et fermement. Ensuite, cet article laisse penser que le statut de la fonction publique interdit toute mobilité, toute adaptation. De nombreuses possibilités existent, mais le cadre juridique proposé retient des logiques qui, traditionnellement, n'étaient pas celles des agents publics : elles étendent au secteur public des pratiques et des fonctionnements qui ont fait la preuve de leur injustice et de leur inefficacité dans le secteur privé. En témoigne la possibilité de bénéficier d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé », en vue de sa reconversion professionnelle. À l'heure actuelle, de telles mises à disposition sont possibles, mais seulement auprès d'organismes privés exerçant des missions de service public et uniquement dans le cadre de l'exercice de ces missions. Vider les emplois publics de leur lien indéfectible avec l'intérêt général, tel est, selon nous, l'un des aspects les plus néfastes de l'article 27. Enfin, aucun accompagnement précis n'est établi au profit des agents publics relevant de la fonction publique territoriale, ce qui constitue une limite évidente aux dispositions de l'article 27.

et la fonction publique hospitalière, des dispositifs d'accompagnement des fonctionnaires dont l'emploi est supprimé. Ceux-ci comprennent un accompagnement en termes de ressources humaines- accompagnement personnalisé, accès prioritaire à la formation, congé de transition professionnelle -et des mesures statutaires, telles que la possibilité de mobilités dans le secteur public, avec des priorités pour le fonctionnaire concerné,

dans un autre ministère éventuellement, mais dans le département où il est établi, de manière à préserver sa vie familiale et son ancrage local. Telles sont les raisons qui nous ont conduits à proposer cet article 27. C'est précisément pour permettre le maintien dans son territoire de vie d'un agent public de l'État dont le poste est supprimé et à condition qu'il accepte d'aller dans un autre ministère que nous prévoyons le congé de transition professionnelle de manière à faire en sorte que cet agent soit formé à un nouveau métier. Il va sans

d'où la modification prévue par le présent projet de loi visant à intégrer cette priorité de mutation dans un cadre plus collectif et plus effectif avec, notamment, la reconnaissance de pouvoirs renforcés au préfet pour favoriser le reclassement d'agents au niveau local, ainsi que je l'ai l'expliqué précédemment. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer les priorités d'affectation ou de détachement pour les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé hors cas de restructuration. Ces deux priorités existent actuellement et ont été supprimées dans le cadre du projet de loi initial. Un amendement de la commission les a réintroduites dans le texte de la commission, afin que les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé hors cas de restructuration puissent en bénéficier. En effet, le dispositif d'accompagnement mis en place par l'article 27 s'applique aux fonctionnaires de l'État dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration.

avons voulu sensibiliser aussi bien la Haute Assemblée que le Gouvernement sur la situation singulière et difficile de deux pays, la Guadeloupe et la Martinique,

vers ladite France métropolitaine pour y travailler. C'était plus facile de mettre la poussière sous le tapis plutôt que de décider de mettre en place des politiques audacieuses et déterminées en matière de développement.

que nous méritons un traitement particulier, qui devrait être inscrit dans la loi, de la même manière que ces migrations forcées l'avaient été. Rien, rien n'a trouvé grâce à vos yeux Pas le moindre amendement ! Et, bien sûr, je ne m'étonne pas du sort qui sera réservé à ce énième amendement portant sur l'article 27.

Alors, je formule encore ma demande, tout en étant très résignée à entendre une réponse commission ? L'article 27 prévoit que les priorités d'affectation des fonctionnaires dont le poste est supprimé dans le cadre d'une restructuration prévalent sur celles qui sont notamment accordées aux fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux en outre-mer. amendement tend à donner aux fonctionnaires originaires d'outre-mer une priorité non seulement sur les fonctionnaires dont le poste est supprimé, mais aussi sur les fonctionnaires qui sont séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, sur les fonctionnaires en situation de handicap et sur ceux qui exercent dans des quartiers difficiles. comprend les attentes des fonctionnaires ultramarins, mais cet amendement pose un problème d'égalité vis-à-vis des autres fonctionnaires qui bénéficient d'une priorité de mutation. Nous avons déjà soulevé ce problème d'égalité lors de l'examen d'un amendement similaire à l'article 11 du projet de loi. D'ailleurs, ma chère collègue, c'est

la ministre nous a elle-même dit que nous pouvions voter le texte en l'état, puisqu'elle ne l'appliquerait pas. Cela me semble une raison suffisante pour rejeter l'article

de transfert d'activité vers une personne morale de droit privé ou de droit public gérant un service public industriel et commercial. Le dispositif de cet alinéa fait l'objet d'une controverse qui n'a échappé à personne. En effet, le mouvement sportif y voit un moyen détourné pour le Gouvernement de forcer le détachement automatique des conseillers techniques sportifs auprès des fédérations. Par ailleurs, les acteurs du monde sportif se sentent trahis par le Gouvernement, car l'alinéa en question a été adopté, comme ma collègue vient de le préciser, alors même que des discussions avaient commencé au sujet de l'avenir des CTS entre les fédérations, les syndicats et le ministère des sports. La ministre des sports, au vu de la polémique suscitée par l'alinéa 11, a promis qu'elle n'appliquerait pas cette disposition aux CTS. Toutefois, nous estimons au Sénat que cette promesse orale n'est pas suffisante. Nous ne mettons pas en cause l'honnêteté de la ministre, mais sa promesse n'engage qu'elle-même. Comment s'assurer que le détachement d'office, s'il est inscrit dans la loi, ne s'appliquera pas aux CTS à l'avenir ? J'entends par avance l'argument du Gouvernement selon lequel l'alinéa 11 vise non seulement les CTS, mais aussi d'autres professionnels, notamment ceux qui exercent dans le cadre des maisons de services au public dont la gestion est confiée à des mutuelles.

pas aux CTS. Mon amendement a pour objet de rétablir un climat propice à une discussion apaisée, de redonner confiance aux acteurs du monde sportif, afin que des négociations sereines sur l'avenir des CTS soient ouvertes. En effet, si l'application de l'alinéa 11 aux CTS en l'absence de concertation préalable n'est pas souhaitable, le ne l'est pas davantage. Les questions du nombre de CTS, de leur formation, de leur répartition au sein des fédérations et de leurs missions doivent être débattues et tranchées. Il ne faudrait pas non plus oublier le cas des conseillers d'animation sportive et des formateurs. Le Gouvernement prévoit une grande loi relative au sport pour le premier trimestre 2020. Fixons-nous cette échéance, monsieur le secrétaire d'État, pour permettre à votre collègue, la ministre des sports, de trouver un accord et d'intégrer dans cette future loi la nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement des CTS.

D'où les pétitions, les manifestations et un mouvement social émanant de concitoyens qui ne sont pas véritablement rebelles ou revendicatifs d'habitude. Ce mécontentement va de la base au sommet, tout simplement parce que les CTS

prioritairement affectés à la montée en puissance du SNU, le service national universel. Que restera-t-il alors des missions traditionnellement exercées par ces agents de l'État ? Et n'oublions pas l'enjeu financier. En effet, les fédérations n'ont pas les moyens

Enfin, quelle contradiction par rapport aux ambitions affichées, c'est-à-dire 80 médailles aux jeux Olympiques de 2024 ! On commence par déstabiliser la préparation olympique, puisque ces CTS ont une véritable épée de Damoclès au-dessus de leur tête, en particulier au moment de la préparation des jeux Olympiques de Tokyo de 2020.

! L'article 28 crée une procédure de détachement d'office pour les fonctionnaires dont le service ou les missions sont externalisés, c'est-à-dire privatisés. Il est symptomatique du désengagement de l'État, dans le droit fil du rapport CAP 2022 et des circulaires récentes du Premier ministre qui encouragent le délestage de missions de l'État sur le secteur privé ou les collectivités. La logique est toujours la même : on asphyxie d'abord le service public. Ainsi, il perd sans cesse du terrain face aux intérêts privés par l'intermédiaire de privatisations successives, de délégations de service public et autres partenariats public-privé. autant de secteurs d'activité dans lesquels les intérêts privés prennent la relève. Quels sont les résultats de ces politiques pour les usagers ? Partout où le service public a perdu du terrain, les tarifs ont augmenté et le service s'est dégradé. Cet article est en définitive l'un des rouages du vaste programme de réorganisation de l'État et des collectivités territoriales, qui contribue à planifier votre suppression de 120 000 fonctionnaires, Ce sont autant de mesures autoritaires contraignantes qui portent un coup à notre fonction publique historique, à la fonction publique « à la française ». Vous avez une conception rabougrie de l'intérêt général, qui se rétrécit à mesure que l'austérité budgétaire progresse à tous les niveaux. C'est bien dans ce cadre-là que s'inscrit ce fait problématique : la perte de statut des agents par le biais de ce détachement automatique et leur éventuelle radiation d'office, à leur demande. Autant dire que les pressions vont être fortes

Ce sont des pans entiers, à l'instar de ces agents, qui pourraient être détachés contre leur gré, sans droit d'option en cas d'externalisation de leur activité vers le privé. À nos yeux, un fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser ou non d'être détaché auprès d'une personne morale de droit privé en cas d'externalisation de son emploi. Le contraindre au détachement revient à nier les principes fondamentaux sur lesquels repose notre fonction publique, qui est une fonction publique de carrière, sujet sur lequel nous revenons depuis le début de l'examen de ce projet de loi. Le Gouvernement justifie cet article par l'existence de situations spécifiques au sein de certaines collectivités qui externalisent des services. Il convenait plutôt de restreindre ce dispositif à ces quelques situations particulières,

opportun de rester parmi les salariés de l'employeur privé, il a la possibilité de démissionner en bénéficiant de l'indemnité de départ volontaire. Ce système beaucoup plus protecteur que le détachement volontaire qui existe jusqu'à présent a été créé à dessein.